et être en mesure de répondre davantage à la forte demande de logements à prix abordable, cet amendement tend à pondérer l'artificialisation résultant de projets de construction de logements sociaux. Il s'agirait des opérations de construction ou d'aménagement destinées à la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements sociaux. Nous souhaitons concilier la mise en oeuvre de l'objectif ZAN, sur lequel nous ne revenons pas, avec la production soutenue de logements sociaux, pour répondre aux 2,4 Il est proposé que cette pondération s'applique sur la première tranche 2021-2031. Un bilan de son application serait réalisé en 2031, permettrait à la conférence régionale de gouvernance du ZAN de faire des propositions pour les étapes décennales ultérieures. La conférence pourrait ainsi vérifier la pertinence de cette mesure au regard des besoins fonciers constatés pour répondre aux enjeux de production de logement, de mixité sociale et fonctionnelle, et d'équilibre entre les territoires. Il est bien précisé que cette pondération constitue non pas une dérogation à l'objectif ZAN, mais un outil facilitateur à utiliser à l'intérieur de l'enveloppe régionale. Quel est l'avis de la commission spéciale ?

Longeot. Cet amendement de Michel Canévet vise à soustraire de la consommation foncière locale les constructions d'équipements de services publics essentiels.

Au rythme fixé par les objectifs du ZAN, 175 000 hectares supplémentaires auront été artificialisés d'ici à 2050, soit 0,3 % de la surface métropolitaine, qui s'étend sur 55 millions d'hectares.

dont au moins 90 % de la superficie est constituée d'espaces naturels ou de zones agricoles, des obligations de zéro artificialisation nette. Ces petites communes constituent l'essence même de la ruralité. Alors qu'elles ont faiblement artificialisé leur territoire, parfois à moins de 2 % ou 3

attendu et légitime. Ce message, c'est notre refus de voir le ZAN congeler le développement de milliers de communes rurales. Ce dispositif ne doit pas condamner nos concitoyens ruraux à l'hibernation, les transformant en Hibernatus que l'on ne réveillerait que pour payer leurs impôts. Le ZAN ne peut pas punir les 10 800 communes vertueuses en matière foncière, qui ont consommé moins de un hectare en dix ans et qui craignent d'être désormais privées de tout droit à construire.

pourquoi on les prive du droit à construire une ou deux habitations au motif de la lutte contre l'étalement urbain. L'inscription dans la loi de la garantie rurale, soit un hectare de surface minimale de développement communal, est donc une condition indispensable à l'acceptabilité du ZAN dans nos campagnes.

comme aux entités les plus grandes, les plus puissantes : communes, villes, intercommunalités, régions ou territoires de Scot. Moins artificialiser le pays ne signifie pas dévitaliser la ruralité, bien au contraire

le tourisme est en plein essor, des entreprises internationales y prospèrent, des start-up s'y installent, le territoire bruisse d'initiatives qui ne demandent qu'à se développer. Nous avons de l'espace, une qualité de vie empreinte de sérénité et de convivialité, des paysages magnifiques ... En somme, c'est un territoire où il fait bon vivre. Il faut vivre dans le Lot ! Nous ne pouvons nous résoudre à devenir une sorte de réserve d'Indiens sacrifiés sur l'autel du ZAN, au prétexte que notre territoire capte du carbone

Elle définit en effet concrètement le potentiel d'artificialisation et, partant, de construction et d'urbanisation dont disposeront les élus locaux dans la décennie à venir, dans la perspective d'atteindre le ZAN d'ici à 2050. L'enjeu principal est bien celui-ci

La capacité d'aménagement de nos collectivités territoriales doit être maintenue. Il s'agit non pas de ne plus faire, mais de faire autrement. Je pense singulièrement aux territoires ruraux, qui ont bien sûr droit au développement- ce droit doit être impérativement protégé et consacré. Il n'est pas question de sacrifier les communes rurales et leurs habitants et de les priver de toute perspective d'aménagement. Toutefois, la solidarité foncière que met en oeuvre cet article, ce fameux hectare

par exemple, de la réalisation d'un projet de territoire. Quoi qu'il en soit, il est évident que les collectivités auront besoin d'être accompagnées par l'État en matière d'ingénierie. En résumé, cette proposition de loi ne fait rien de moins qu'esquisser le visage futur de la France. Il s'agit d'un pas essentiel vers la transformation

C'est une façon de consacrer notre volonté, si souvent affirmée dans cet hémicycle, de reconnaître les spécificités des zones rurales, par une équitable répartition de l'effort attendu en matière de réduction de l'artificialisation. Cette mesure corrige

à la bétonisation générale des grandes métropoles, ce serait alors la double peine. J'ajoute que le rapporteur Jean-Baptiste Blanc a largement fait justice de la fable selon laquelle cette mesure viendrait réduire de manière drastique l'enveloppe d'artificialisation. En effet, retenir comme critère un pourcentage de la surface urbanisée

Une garantie rurale définie sur la base d'un hectare par commune représenterait 29 % de cette enveloppe. Cela réduirait d'autant les possibilités des territoires en tension, qui accueillent une population nombreuse, ainsi que des activités économiques, sans permettre d'atteindre collectivement les objectifs fixés par la loi Climat et résilience.

Cette solidarité territoriale doit se traduire dans la planification. Dans le cadre du dialogue intercommunal et afin de tenir compte des besoins futurs de développement des communes rurales, nous proposons donc de créer une « enveloppe territoriale de solidarité foncière », qui aura pour objet de conserver, à l'échelle intercommunale, quelques hectares non territorialisés pour anticiper les projets encore inconnus au moment de l'approbation du document. Cette enveloppe pourrait être utilisée uniquement si le projet proposé par une commune peut être justifié par un manque de foncier et si aucune solution de renouvellement urbain n'est possible. À titre d'exemple, une intercommunalité disposant d'une enveloppe de cent hectares à consommer dans les Enaf pourrait décider de créer une réserve de trois hectares

cet article, de manière à éviter des situations locales particulièrement préjudiciables aux territoires ruraux, à l'avenir de l'agriculture et, évidemment, à la souveraineté alimentaire que nous défendons tous. En effet, d'une part, les communes pourraient se trouver dans l'impossibilité d'installer de jeunes agriculteurs d'autre part, les maires pourraient se voir contraints de choisir entre la construction d'une habitation et celle d'un bâtiment agricole, question évidemment complexe. Enfin, rappelons que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation commercialisation des produits agricoles, ainsi qu'au stockage et à l'entretien du matériel constituent déjà des dérogations au droit commun de l'urbanisme, dans la mesure où ce type de constructions et d'installations est autorisé en dehors des espaces urbanisés de la commune, dans le cadre du règlement national d'urbanisme,

c'est en quelque sorte récompenser les gros consommateurs de foncier d'hier. Plutôt que de corriger les effets de bord de l'application du ZAN, on les renforcera ! Eh oui ! Bien sûr ! En outre, ce critère ne prend nullement en considération les dynamiques démographiques, d'emploi, ou de développement. Son seul avantage, aux yeux du Gouvernement, est d'offrir une garantie plus limitée en volume. Je rappelle aussi qu'il n'existe pas, à ce jour, de données fiables

de celles-ci, sans parler de ce passage extraordinaire du rapport qui indique que « la taille des petites communes est devenue un handicap lorsque l'acte I de la décentralisation a supprimé la tutelle préfectorale et leur a confié de nouvelles compétences, notamment en matière d'urbanisme »,

pénalise les communes qui n'ont que très peu artificialisé. De nombreuses communes rurales où l'on avait peu construit redeviennent attractives grâce non seulement au télétravail et à la fibre, mais aussi en raison de la qualité de vie ; elles risquent d'être trop lourdement pénalisées par l'objectif fixé. La surface artificialisée est de 7,9 % à l'échelon national. Nous proposons que les communes dont le taux d'artificialisation est inférieur à 3 % puissent bénéficier d'un hectare supplémentaire à construire pour les dix années à venir.

M. Bernard Fialaire. L'article 7 confère un droit à l'hectare à toutes les communes, sans faire de distinction. Les élus chargés de l'élaboration des Scot n'ont pas l'intention d'interdire tout droit au développement aux communes rurales.

30 % de l'enveloppe de cette décennie serait ainsi mobilisée par ce droit à l'hectare. Le présent amendement vise donc à préserver une définition plus souple de la surface minimale de développement communal, en supprimant la référence à l'hectare dans le cadre des Scot.

n'a jamais été aussi alarmant. La politique de l'urbanisme joue un rôle important en la matière en participant à la préservation des milieux naturels et à la protection de la biodiversité. Pour ce faire, les collectivités territoriales territoriales doivent inscrire dans le schéma de cohérence territoriale leurs orientations et les modalités de leurs actions en matière de préservation de la biodiversité. Dans le cadre des plans locaux d'urbanisme, il est prévu seulement qu'elles dans le plan d'aménagement et de développement durable, les orientations des politiques de maintien ou de remise en état des continuités écologiques. Le présent amendement vise, dans un premier temps, l'inscription de la politique de préservation de la biodiversité dans les plans

Cet amendement vise à prendre en compte les objectifs de la politique énergétique et de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets dans le calcul du taux d'artificialisation contexte d'urgence climatique, il est essentiel de favoriser le développement de projets qui contribuent à la transition écologique locale, afin de poursuivre et d'accompagner les efforts engagés par les territoires en la matière, tout en respectant les objectifs de « zéro C'est particulièrement le cas des activités de gestion des déchets et de production d'énergies renouvelables. Compte tenu de l'importance de ces projets dans la mise en oeuvre de la transition écologique de nos territoires, et en parfaite cohérence avec les objectifs de la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

! Il se trouve qu'il faut encourager- et je suis mille fois pour ! -l'économie circulaire, les énergies renouvelables, mais tout cela sans consommer de terrain

L'amendement vise à clarifier le statut des friches, qui est incertain en l'état actuel du droit, en précisant que celles-ci doivent être regardées comme des surfaces artificialisées au sens de la stratégie de sobriété foncière et de lutte contre l'artificialisation des sols. Cette disposition permettrait de favoriser la réhabilitation et le recyclage foncier des friches commerciales, artisanales ou industrielles. La réutilisation d'emprises foncières enfrichées n'entraînera aucune consommation d'espace ni d'artificialisation au sens de la loi Climat et résilience. À l'inverse, leur renaturation améliorerait le solde net d'artificialisation de la collectivité. que nous proposons est conforme à l'esprit de l'objectif ZAN, qui repose sur l'utilisation prioritaire de friches et de terrains déjà artificialisés ou situés dans un périmètre urbain, dans une logique de densification et de limitation de l'étalement urbain.

Arnaud. Les jardins particuliers, potagers ou d'agrément constituent des espaces verts propices à la biodiversité et participent ainsi aux objectifs nationaux et internationaux en matière de climat et de protection de la biodiversité.

elles ne devront faire l'objet d'aucun traitement contenant des produits phytosanitaires. En effet, les intrants sont une des causes principales de baisse de la biodiversité. Sans les animaux, le vivant, la nature

À la grande loterie de la valse des continents et des climats, la France a tiré le gros lot. Trois bonnes fées se sont penchées sur son berceau : la fée Géologie, la fée Géographie et la fée Biodiversité. Elles lui ont offert, rassemblée dans un mouchoir de poche, une extraordinaire diversité de paysages.

un enjeu de souveraineté. Il est ainsi proposé que les surfaces nécessaires à la construction de nouvelles scieries et autres équipements sylvicoles dans notre pays ne soient pas décomptées au titre du ZAN.

En vertu des dispositions de la loi Climat et résilience du mois d'août 2021, les bâtiments agricoles seront considérés comme des surfaces artificialisées à partir de 2031. Dans un contexte de sobriété foncière, cette disposition ne manquera pas de soulever de nombreuses difficultés et soumettra les élus locaux à des dilemmes en matière d'aménagement. Les maires pourraient devoir choisir entre la construction d'habitations et le développement ou la création d'exploitations agricoles. rappelons que les entreprises agricoles, socles non délocalisables de l'économie des territoires ruraux, auront à répondre au cours des prochaines années aux obligations de mise aux normes pour le bien-être animal, entraînant l'extension éventuelle des bâtiments existants. Les exploitations agricoles devront également s'adapter aux enjeux climatiques, ce qui supposera des infrastructures nouvelles pour la préservation de leur production et leur diversification. Les emprises artificialisées nécessaires à l'exploitation agricole constituent déjà des dérogations au droit commun de l'urbanisme, dans la mesure où ce type de constructions et d'installations est autorisé

conçues pour affronter les aléas climatiques et pour assurer la souveraineté alimentaire de notre pays. Il s'agit de préciser qu'une surface occupée par des constructions, installations et aménagements nécessaires à l'exploitation agricole sera considérée comme non artificialisée. Notre objectif est de donner aux jeunes l'envie de s'installer et des perspectives de développer durablement une activité agricole. Dans le prolongement de nos échanges en commission, nous souhaitons aussi aborder ce sujet essentiel qu'est l'avenir des exploitations agricoles, notamment éclaircir le changement de destination des bâtiments agricoles. Sans création de surfaces nouvelles, une réhabilitation ne doit pas être considérée comme une nouvelle artificialisation. L'objectif est bien de favoriser la réappropriation du bâti existant pour, par exemple, répondre à des besoins en logement ou créer de nouvelles activités dans les territoires ruraux. Il existe en effet, sur nos territoires, des centaines de granges, de bâtiments d'élevage ou encore de bâtiments

de loi prévoit explicitement que les surfaces végétalisées à usage résidentiel, secondaire ou tertiaire- jardins particuliers, parcs, pelouses -soient considérées comme non artificialisées. artificialisées. L'article L. 151-23 du code de l'urbanisme prévoit, quant à lui, l'identification d'espaces à protéger pour des considérations écologiques dans les zonages des plans locaux d'urbanisme, notamment les trames vertes et bleues. Ce sont des zones inconstructibles, mais elles peuvent être intégrées dans un zonage à urbaniser ou une zone urbaine. Aussi, afin de ne pas pénaliser le développement des communes qui s'engagent dans la création d'espaces protégés, nous proposons par cet amendement de considérer ces espaces comme non artificialisés. Dès lors, ils ne doivent pas être retenus dans l'assiette déterminant les futurs droits à construire.

Mme Maryse Carrère. Dans la série des exclusions de la nomenclature, cet amendement vise à considérer comme non artificialisées les surfaces occupées par des ouvrages de stockage temporaire des eaux, comme les bassins tampons ou les bassins d'orage. L'amendement n° 173, présenté par M.

et l'estimation du coût des opérations de renaturation. En effet, indépendamment de leur nature, les friches ne sont aujourd'hui qu'imparfaitement recensées. Entre rareté du foncier et lutte contre l'artificialisation des sols, la reconversion des espaces constitue pourtant un véritable enjeu dans la mise en oeuvre de l'objectif ZAN, reposant sur une logique de réduction de l'artificialisation nette des sols. Les opérations de renaturation produiront donc des droits nouveaux à artificialiser.

dans un état annexé à leurs documents d'urbanisme, en particulier lors de la révision de ces documents, les friches potentiellement mobilisables situées sur leur territoire. Ce travail pourrait, par exemple, être mené par des bureaux d'études, qui sont déjà compétents en la matière. Notre objectif est que le potentiel de revalorisation de ces terrains puisse être plus facilement identifié,

n° 209 rectifié. L'article 9 permet de délimiter des périmètres de densification et de recyclage du foncier dans lesquels l'utilisation des espaces végétalisés ne sera pas prise en compte pour évaluer l'atteinte des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols. Or, le calibrage de la trajectoire d'artificialisation conditionnant l'enveloppe de renaturation nécessaire à la mise en oeuvre de la stratégie territoriale se fera à l'échelle du Scot. le présent amendement, il est donc proposé que des espaces préférentiels de densification, ainsi que leur volume soient identifiés dans le Scot, en articulation avec la trame verte et bleue du territoire. parole est à M. Bernard Fialaire. L'article 9 prévoit que toutes les surfaces végétalisées à usage résidentiel, de loisirs, ou d'infrastructures de transport soient considérées comme non artificialisées. non artificialisées. Si cette évolution permet de répondre aux nombreuses inquiétudes quant à la comptabilisation de l'artificialisation des projets en extension urbaine, elle obère très fortement la capacité de densification dans l'enveloppe urbaine existante et va à l'encontre du principe visant à « refaire la ville sur la ville ». L'introduction de périmètres de densification et de recyclage foncier par les communes et EPCI constitue une contrepartie pour permettre les projets de densification. Afin de favoriser davantage le recyclage urbain, il est donc proposé d'intégrer les friches aux périmètres pouvant être définis par les EPCI aux termes des modifications apportées au texte par la commission.

c'est cela, la logique du ZAN. En revanche, en faisant entrer les parcelles privées des lotissements dans la nomenclature à partir de 2030, on va grignoter l'espace agricole,

Je vous propose de prolonger notre séance afin d'achever l'examen de ce texte. Il nous reste cinquante-trois amendements à examiner

Les dispositions de cet article qui visent à décompter de l'artificialisation constatée sur la période les terrains « perdus à la mer » du fait du recul du trait de côte, c'est-à-dire rendus inutilisables,

cent ans ! Plus précisément, pour la commune de Gouville-sur-Mer, les surfaces urbanisables sont évaluées à moins de quatre hectares pour la période 2021-2031, alors que nous devons relocaliser sept à huit hectares d'infrastructures touristiques dans le cadre du projet partenarial d'aménagement Vous imaginez bien que, sans ce décompte, le seul effort de relocalisation grèverait toute possibilité de développement. Face à l'érosion côtière, que nous ne contrôlons évidemment